La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 janvier 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. est adopté. Par lettre en date du 9 janvier, le Gouvernement demande l'inscription des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire à l'ordre du jour du jeudi 30 janvier, à

la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

des réserves sur l'arrêt de projet, ce qui soulève des inquiétudes. Il n'est en aucun cas question de remettre en cause les observations formulées sur la bande des 100 mètres ou sur les zones proches du rivage, dont la protection est légitime et tout à fait souhaitée.

et a émis un avis favorable, assorti d'observations. Ces dernières ne constituent nullement une remise en cause du caractère urbain de plusieurs des secteurs, comme vous l'évoquez. Elles visent à renforcer la sécurité juridique du PLUI, notamment au regard des évolutions récentes apportées à la loi Littoral (schéma de cohérence territoriale) applicable sur la zone depuis 2014. Ainsi, lors de l'examen du projet arrêté, l'État a constaté que la communauté avait retenu une qualification différente du SCOT pour certains secteurs, à savoir celle de village. Ces observations visaient donc simplement à répondre à l'exigence de compatibilité du PLUI arrêté avec le SCOT en vigueur. Un autre point d'achoppement portait sur la qualification de certains secteurs en zones urbaines dans une période transitoire au cours de laquelle cette qualification n'a pas encore été confirmée dans le SCOT. Après examen, il semble que le zonage urbain de ces secteurs ne soit pas remis en cause par l'avis de l'État. C'est un point important, parce que ce zonage ouvre la possibilité de délivrer, sous réserve de l'accord du préfet, des autorisations de construire. Les règles de constructibilité prévues par le projet de PLUI pour ces secteurs ne répondaient pas tout à fait à ce qu'autorise la loi ÉLAN. Des ajustements étaient donc nécessaires.

j'appelle votre attention sur le déploiement des maisons France services (MFS), annoncé par le Premier ministre le 4 mai dernier. Il existe aujourd'hui 1 340 maisons de services au public (MSAP). Avec l'annonce du Premier ministre, 500 maisons France services vont être mises en place-

La Cour des comptes souligne, dans son rapport de mars 2019, le risque pour les MSAP de devenir « des structures de délestage de l'État et des opérateurs qui y verraient l'occasion de réduire leurs coûts de réseaux en les transférant aux collectivités ». Autrement dit, une charge financière supplémentaire pour les territoires. De plus, elle dénonce « l'impasse du financement des MSAP », dont les fonds, qui reposent pour moitié sur les collectivités, ne seraient « pas de nature à en garantir la pérennité

Je pense également aux MSAP d'Albestroff, de Dabo et de Lorquin, toujours en Moselle. Que vont-elles devenir ? Devront-elles fermer ? Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, quel sera l'avenir des MSAP. Que compte faire le Gouvernement pour compenser et réparer le préjudice financier des communes qui ont déjà investi dans ces structures ? Par ailleurs, pouvez-vous nous dire comment vous allez aider les communes à financer ces maisons France services, notamment dans les zones rurales ? La parole est à Mme la ministre.

la structure d'Entrange, qui répondait aux trente critères de qualité de service, a été labellisée. Un nouvel audit va être effectué dans les prochaines semaines pour les structures de Boulay-Moselle

doivent être théoriquement ouvertes. Elles ont été créées pour répondre aux besoins des Français dans leurs démarches administratives, principalement en zones rurales et périurbaines, périurbaines, afin de conserver un lien physique avec un certain nombre d'organismes et de services de l'État. Ces nouvelles structures labellisées seront ouvertes au moins cinq jours par semaine et chacune d'entre elles devra disposer de deux personnes formées à l'accueil du public, capables d'apporter une aide dans les démarches. Or les collectivités locales s'inquiètent de leur financement. Les préfets ont dû fournir la liste des maisons de services au public existantes

pour recevoir le public ? Que compte faire le Gouvernement pour le réseau actuel de maisons de services au public non labellisées et éviter qu'elles ne ferment ? Il s'agit de pérenniser ces emplois sur nos territoires.

Pour répondre à votre question, les MSAP qui n'ont pas été labellisées seront accompagnées financièrement jusqu'au 31 décembre 2021.

par exemple, qui émane de la Caisse des dépôts et consignations, investit ainsi 30 millions d'euros pour assurer le déploiement de France services. Sur cette enveloppe, 17 millions sont alloués à La Poste, 10 millions à l'animation globale du réseau et 3 millions d'euros permettront le déploiement de structures France services mobiles. L'État apporte un soutien financier aux structures France services labellisées, ainsi qu'aux MSAP en cours de montée en gamme : sa participation aux dépenses de fonctionnement de la structure consiste en un forfait de 30 000 euros, contre 25 000 euros par an en moyenne aujourd'hui. L'État accompagne également les collectivités dans leur investissement au travers

territoriales. Madame la ministre, en créant l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) afin de remédier aux disparités constatées dans notre pays, le Gouvernement a souhaité améliorer la cohésion territoriale. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L'article 3 de la loi du 22 juillet 2019 portant création de cette agence spécifie que « le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins Pourtant, à la lecture du décret du 18 novembre 2019 relatif à cette agence, il s'avère qu'aucun représentant spécifique du littoral n'a été identifié. Ce sont tous les territoires littoraux de la France hexagonale et des outre-mer, reconnus par la loi Littoral de 1986 pour leur spécificité et le caractère exceptionnel de leur richesse en biodiversité, qui sont ici oubliés. Je ne peux m'y résoudre en tant que sénateur d'un département disposant d'une frange littorale importante et président de l'Association nationale des élus du littoral. En parallèle, plusieurs associations d'élus bénéficient d'un siège, notamment l'Association nationale des élus de la montagne. Une telle : si les spécificités de la montagne sont prises en compte, pourquoi celles du littoral ne le sont-elles pas ? Submersion marine, érosion côtière, changement climatique, biodiversité, préservation du patrimoine, économie bleue ... Ces sujets ne méritent-ils pas d'être pleinement considérés dans le cadre d'une telle agence ? Après plusieurs courriers vous alertant sur ce sujet, dont un émanant de députés de votre majorité, et une tribune signée par plus de 140 parlementaires, la situation n'a malheureusement pas évolué. Pour une cohésion nationale forte, qui vous est chère, madame la ministre, et dans l'intérêt des 6 millions d'habitants résidant sur nos littoraux, ce décret doit être modifié. Une révision indispensable pour redonner au littoral, ainsi qu'à ses nombreux acteurs, la juste place qu'ils doivent naturellement avoir. Quelles sont donc vos intentions à ce sujet ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s'est réuni pour la première fois le jeudi 12 décembre 2019, est composé de manière à concilier deux impératifs presque antagonistes : une taille réduite et pilotable, d'une part ;

les élus locaux s'interrogent sur la portée des modifications de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issues de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. » Les élus locaux s'interrogent sur le caractère obligatoire de procéder le même jour, et lors de la même séance, à l'élection du président de l'EPCI, des vice-présidents et des autres membres du bureau. En effet, les métropoles comportent un nombre important d'élus et leurs représentants ne sont connus qu'à l'issue du deuxième tour des élections municipales. À l'échelle d'une métropole, il est donc difficile d'organiser une gouvernance en amont du résultat des élections municipales, contrairement à ce qui peut être fait à l'échelle d'une commune. il est de pratique courante, au sein des métropoles, de procéder, dans un premier temps, à l'élection du président puis, dans un second temps, lors d'une autre séance- généralement une quinzaine de jours après -, à l'élection des vice-présidents et du bureau. La modification de l'article L. 5211-6 du CGCT a eu pour finalité de rendre obligatoire la lecture de la charte de l'élu local lors de l'élection du président et des vice-présidents de l'EPCI. Peut-on considérer que les dispositions de cet article sont respectées si l'élection du président et des vice-présidents a lieu lors de deux séances distinctes, mais que la charte de l'élu local est lue par le président lors de chacune de ces séances ?

Monsieur le sénateur Dany Wattebled, l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : « Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local [ ...] » Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 31 mars 2015 pour intégrer la lecture de la charte de l'élu local après l'élection de l'exécutif intercommunal. L'intention du législateur était de mettre en oeuvre la proposition n°°24 du rapport de la mission d'information sur le statut de l'élu, en créant une charte de l'élu local comme cadre déontologique. Lors des débats parlementaires en commission des lois, le rapporteur avait précisé que les conseils municipaux et les conseils communautaires seraient concernés de la même façon par cette disposition. Je vous confirme ainsi que, après le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2020, le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau d'un EPCI à fiscalité propre seront élus lors de la même réunion du conseil communautaire. J'attire votre attention sur le fait que la disposition prévoyant que, « après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires » demeure au sein de l'article L. 5211-6 du CGCT. Cette disposition permet de laisser un temps d'échange aux élus des conseils communautaires pour procéder à l'élection de leurs exécutifs. Dès lors, en prévoyant un délai de près de cinq semaines entre l'élection des conseillers communautaires et l'élection de leurs président, vice-présidents et membres du bureau, le législateur a reconnu la nécessité, pour les EPCI à fiscalité propre, de bénéficier d'un temps plus plus long pour constituer leurs exécutifs. Par comparaison, l'article L. 2121-7 du CGCT ne laisse qu'une semaine aux conseils municipaux pour procéder à l'élection des maires et des adjoints. Il reste enfin loisible, de façon concrète, tout en organisant l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau dans la continuité de celle du président et lors de la même réunion, de réserver une suspension de séance dans le déroulement de ces scrutins. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur l'importance du trafic poids lourds, plus particulièrement celui en transit sur la RN10 entre Poitiers et Bordeaux. poids lourds ne respectent ni les distances de sécurité, ni l'interdiction de doubler, ni la limitation de vitesse, au point que les routiers eux-mêmes disent prendre un risque pour leur vie et celle des automobilistes. À l'insécurité routière s'ajoutent la pollution sonore ainsi que la pollution de l'air et des sols, si bien que les agriculteurs, soucieux de produire de la qualité,

Au regard des conséquences de ce trafic sans cesse grandissant en termes de sécurité routière, sanitaire, environnementale, sociale et économique, sans oublier le coût d'entretien de la chaussée et la mobilisation des forces de l'ordre, plus de 7 000 personnes ont signé une pétition citoyenne demandant que les poids lourds

qu'« il fallait se préoccuper des poids lourds en transit pour faire en sorte qu'ils n'aient pas la tentation d'emprunter des itinéraires gratuits ». Ma question est simple : que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'État, pour régler ce problème ?

complète sur la route nationale 10 entre Poitiers et Bordeaux du trafic de poids lourds serait contraire au principe de libre circulation des marchandises sur le réseau structurant national. Vous le savez, la jurisprudence du Conseil d'État est constante sur ce point, afin de garantir un principe fort de la réglementation européenne. Pour autant, les services de l'État chargés du contrôle sont mobilisés sur le terrain pour assurer le respect des réglementations applicables au transport routier, afin de prévenir les risques de surcharge. Il le temps de conduite et de repos des chauffeurs, ainsi que le respect de leurs conditions de travail. Le Gouvernement entend donc prendre des mesures d'amélioration des infrastructures. Une telle politique est mise en oeuvre sans porter préjudice aux concertations qui pourraient intervenir à l'avenir. De nombreuses opérations de sécurisation de cet axe ont d'ores et déjà été engagées : la mise en service de la 2x2 voies entre Reignac et Chevanceaux ; l'étude du remplacement de six carrefours dans la Vienne par des échangeurs dénivelés avec mise à 2x2 voies dans le secteur de Croutelle ; l'étude de la suppression des derniers carrefours en Charente, notamment sur la commune de Mansle ; le diagnostic de sécurité sur la rocade d'Angoulême, en vue d'améliorer, dès 2020, les modalités d'information des usagers de la route, en particulier sur les congestions récurrentes et les risques d'accidents ; enfin, le diagnostic de sécurité sur la section entre Virsac et Angoulême. Au regard de ces nombreux projets d'amélioration de l'infrastructure routière, le Gouvernement va demander à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de s'assurer que chaque calendrier d'opération soit respecté au mieux. Par ailleurs, le Gouvernement mandatera la préfète de la Charente, afin que des dispositifs de contrôle fixes et mobiles soient déployés de façon privilégiée sur cet axe, de manière à renforcer la répression contre les poids lourds qui ne respecteraient pas les différentes réglementations. La parole est

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question concerne les abus de faiblesse liés à la généralisation de la signature électronique à distance. Ce phénomène est principalement constaté dans le secteur des assurances. En effet, un contrat d'assurance peut être souscrit en quelques minutes par téléphone après la simple expression du consentement. Ce dernier se matérialise généralement par un code reçu par SMS qu'il faut répéter à voix haute au courtier ou encore par une touche de téléphone sur laquelle il faut appuyer. Nous en conviendrons tous, cette spécificité accordée aux assurances est pratique lorsqu'il s'agit d'assurer dans l'urgence sa nouvelle voiture. Mais force est de le constater, elle est bien souvent utilisée à mauvais escient. Ce type de vente est souvent expéditif, afin que le client n'ait pas le temps de prendre la mesure de la situation. Les personnes isolées, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées, sont bien souvent démunies face à des professionnels de la vente qui n'hésitent pas user de tous les stratagèmes possibles afin de parvenir au plus vite à la signature d'un contrat aux modalités hasardeuses. Bien souvent, ces personnes ne réalisent pas qu'elles viennent de souscrire à un contrat d'assurance, ce qui rend la tâche des familles qui les accompagnent bien plus difficile que dans le cas d'un simple démarchage, en porte-à-porte. Ainsi, le délai de rétractation de 14 jours n'est souvent pas suffisant pour débusquer la supercherie. Sur la seule année 2018, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé 92 entreprises et en a épinglé 27. Dans la plupart des cas, les démarcheurs recourent à des allégations mensongères, afin de recueillir l'accord verbal du consommateur ou obtenir la signature électronique du contrat. Ma question sera la suivante, madame la secrétaire d'État : au regard des nombreux cas constatés d'arnaques et de ventes forcées, en particulier auprès des personnes âgées ou handicapées, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement concernant la lutte contre ce phénomène inquiétant.

C'est pourquoi le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif et intrusif. Il a ainsi demandé au Conseil national de la consommation (CNC) d'établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités

a nourri les travaux sur ce sujet, en particulier la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Ce texte a fait l'objet d'un premier examen par l'Assemblée nationale le 6 décembre 2018, puis par le Sénat le 21 février 2019.

en nous assurant que l'engagement pris par la profession est clairement respecté. Vous avez raison, madame la sénatrice, il n'est pas légitime qu'un accord sur un sujet aussi complexe qu'un contrat d'assurance soit obtenu sans traçabilité

exploitant des listings commerciaux pour joindre les occupants- principalement les propriétaires -de maisons individuelles qui pourraient bénéficier de travaux d'isolation à 1 euro.

en cause le projet de taxe sur les géants du numérique. Les vins pétillants, dont le champagne, épargnés par les premières sanctions, seraient également concernés, ce qui représente 700 millions d'euros supplémentaires. Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché américain s'est élevé à un milliard d'euros en 2018. Sur les six premiers mois de 2019, les exportations étaient en hausse de 10 % en valeur et de 2 % en volume. Or, depuis bientôt trois mois, la profession enregistre une chute drastique des importations américaines, de l'ordre de 30 % en valeur, sur les vins en bouteilles, par comparaison avec le mois de novembre 2018. Les exportateurs ont réduit leurs marges, mais ils redoutent de perdre des parts de marchés qui seront difficiles à reconquérir, d'autant que ces mesures entraîneront des distorsions de concurrence. Le 16 décembre dernier, lors du Conseil Agriculture et pêche à Bruxelles, le ministre de l'agriculture a demandé à la Commission de renforcer les soutiens à la filière vitivinicole. les mesures proposées vont dans le bon sens, elles demeurent insuffisantes pour faire face aux conséquences directes pour la filière. En conséquence, qu'en est-il de la mise en oeuvre d'un fonds de compensation des mesures d'aides à la promotion ou de la résolution du conflit avec les États-Unis ? Le 6 janvier dernier, M. Bruno Le Maire a une nouvelle fois appelé les États-Unis à la raison. Toutefois, pour l'heure, on ne constate aucun effet. Madame la secrétaire d'État, il y a urgence à agir, afin de ne pas fragiliser l'ensemble de la filière, victime d'un conflit qui ne la concerne pas. La

dans le conflit opposant les États-Unis et l'Union européenne au sujet des subventions accordées à Airbus, l'OMC a tranché et autorisé les États-Unis à appliquer des sanctions à l'encontre de biens européens importés sur leur Dans la mesure où il est vraisemblable que l'OMC sanctionne aussi, dans quelques semaines, les produits américains importés en Europe, pour des subventions accordées à Boeing, l'Union européenne a d'abord tenté de négocier avec les États-Unis, pour éviter une escalade de sanctions qui mette à mal l'économie de nos territoires respectifs.

Pour la France, les produits les plus touchés sont les vins tranquilles en deçà de 14 degrés conditionnés dans des contenants de moins de 2 litres, auxquels est imposée une taxe additionnelle de 25 %. Toutes les régions viticoles françaises sont visées, à hauteur de 306 millions d'euros annuels. Les exportations françaises aux États-Unis des vins taxés ont représenté 25 % de l'ensemble des exportations européennes de vins vers les États-Unis. Pour aider au plus vite la filière, injustement frappée et en difficulté, le Gouvernement a immédiatement mis en oeuvre des mesures de soutien : doublement du budget de la promotion des vins français développés aux États-Unis et dans plusieurs autres pays stratégiques, notamment en Asie, dans le cadre de la concession de service public Sopexa ; renforcement des actions de promotion conduites par Business France, notamment sur les indications géographiques et les appellations d'origine contrôlée ; opérations collectives de promotion à l'export sur 38 marchés à potentiel en 2020 mise en oeuvre de mesures de bienveillance concernant des délais de paiement ou des remises et de l'assurance prospection portée par Bpifrance. Au-delà des mesures nationales, c'est bien sûr au niveau européen que doit se porter le soutien Ainsi, à notre demande, l'Union européenne a déjà accordé diverses mesures de souplesse et de simplification des fonds de promotion. Mais la France, notamment par la voix de Didier Guillaume, continue de solliciter, lors de chaque Conseil européen de l'agriculture,

Je pensais que la fameuse loi Grand âge serait le grand soir des financements. Or je m'aperçois que nous sommes toujours dans les petits matins précaires des renoncements. Les structures d'aides à domicile sont en effet désemparées elles refusent de s'habituer à des effets d'annonces non suivies de résultats dans des délais raisonnables. La situation est pourtant désastreuse et alarmante : alors que 600 millions d'euros sont nécessaires pour rattraper le retard et améliorer un contexte tendu, seuls 50 millions d'euros ont été octroyés en 2019, 50 autres millions étant promis pour 2020, soit deux fois moins que ce qui avait été prévu en 2018. En Lot-et-Garonne, les tarifs horaires appliqués pour les structures d'aide et d'accompagnement à domicile sont toujours fragiles et évidemment non pérennes : 20,73 euros pour un prix de revient de 21 euros. Dans le même temps, les 520 000 euros fléchés en 2019 posent question : le département ne se prononce pas pour 2020, les conditions d'attribution à remplir par le biais des appels à candidatures étant toujours inconnues. Imaginez le désarroi de toutes ces structures et de leur personnel À quand une réforme ambitieuse de la tarification des services d'aide à domicile ? À quand une remise à plat des modèles d'intervention ? À quand un financement à la hauteur des enjeux, alors qu'il faut treize intervenant à domicile pour être rémunéré légèrement au-dessus du SMIC ? Madame la secrétaire d'État, quand pourrons-nous espérer passer des promesses, des commissions et des rapports aux actes réels, responsables et immédiats ?

des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Le financement des SAAD relève de la compétence des conseils départementaux. Le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, pris pour l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, vise à préfigurer un nouveau modèle de financement des SAAD, afin d'assurer l'accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires, permettre une plus grande équité de traitement, de rendre l'offre plus lisible, d'assurer une meilleure transparence tarifaire, et de mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers. Le modèle rénové que nous envisageons repose sur un tarif de référence nationale applicable à tous les SAAD, et un complément de financement appelé « modulation positive

Il appartient aux départements de répartir ces crédits entre les SAAD retenus dans le cadre d'un appel à candidatures et dont le cahier des charges a été précisé dans le décret. Les critères de sélection des candidatures portent notamment sur le profil des personnes prises en charge, l'amplitude horaire d'intervention et les caractéristiques du territoire d'intervention, afin de renforcer l'attractivité des métiers du secteur. La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée aux SAAD à l'issue de l'appel à candidatures relève de la négociation entre le département et les SAAD lors de la signature du CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) ou d'un avenant à ce contrat. Les départements bénéficiaires de ces crédits devaient transmettre à la CNSA les données relatives à l'utilisation des crédits au plus tard le 15 octobre 2019. Concernant les ARS (agences qui pourraient intervenir en faveur des SAAD seraient les financements alloués dans le cadre de l'accompagnement à la constitution d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, regroupant les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile. La parole

a la responsabilité de répondre au souhait de 95 % des Français, qui désirent vivre le plus longtemps chez eux, à domicile. Ne pas les entendre serait ne pas entendre une évolution majeure de notre société.

et de la santé : « Madame la ministre, nous vous alertons régulièrement sur les carences en matière de professionnels de santé dans différents secteurs. On pense évidemment aux déserts médicaux dus au manque de renouvellement des médecins généralistes tant en secteur rural qu'en ville dans les services d'urgence des hôpitaux. On pense aussi à la difficulté d'avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste ou de trouver un médecin traitant. « Je souhaite aujourd'hui vous alerter et attirer votre attention sur le déficit constaté partout en France de candidats aux sessions de formation d'aide-soignant, métier de santé pourtant indispensable dans le dispositif de prise en charge des malades. « En effet, si je me réfère à l'exemple de mon département, il y avait encore récemment en Drôme deux sessions de formation, avec chacune 60 stagiaires qui se dirigeaient ensuite vers le métier d'aide-soignant.

Toutefois, l'évolution du nombre des diplômés est restée quasi stable : il était de 22 800 en 2018. Afin de favoriser l'accès à cette formation et de mieux reconnaître les compétences des aides-soignants dans leur pratique professionnelle, plusieurs actions ont été engagées depuis 2018. Leur mise en oeuvre se poursuit, notamment dans le cadre des Ma santé 2022 et Investir pour l'hôpital. La valorisation de la formation et, par là même, de la profession d'aide-soignant est au coeur des mesures portées par le ministère. Un groupe de travail associant tous les acteurs concernés s'est constitué en avril 2019. Il a engagé une refonte des référentiels métier et formation, et formation, qui est en cours de finalisation en vue d'une mise en place à la rentrée de septembre 2020. La réforme est aussi l'opportunité de mettre en place des passerelles avec d'autres professions et, donc, de décloisonner l'exercice de la profession d'aide-soignant.

La mobilisation continue au niveau des agences régionales de santé (ARS) pour valoriser le métier et desserrer le calendrier des concours existants, qui était trop étalé dans le temps. J'en veux pour preuve qu'il fallait attendre près d'un an entre son inscription au concours et l'entrée dans la formation, ce qui ne permettait pas aux jeunes intéressés par le métier d'aide-soignant de se projeter aussi loin.

Or, depuis cet été, les urgences de Sisteron n'ont jamais rouvert la nuit. Or le bricolage comme la bonne volonté ne sont pas des politiques acceptables, surtout quand la sécurité des patients mais aussi la nécessaire accessibilité aux services publics sur tout le territoire et dans les mêmes conditions sont en jeu. Élu des Alpes-de-Haute-Provence, je ne peux pas accepter d'être le sénateur d'un département où le service public de la santé n'existe que le jour. Je ne peux accepter non plus que, à terme, ce service public de nuit soit assuré dans d'autres départements, ce qui contraindrait les patients à des déplacements encore plus longs, dans des conditions parfois plus difficiles-

Madame la secrétaire d'État, la publication de ce rapport laisse entendre à tous les acteurs de la santé du département que l'hôpital de Sisteron ou d'autres services d'urgence du département, eux aussi fragilisés, pourraient être les premiers concernés par ces fermetures permanentes la nuit. Pourtant, des solutions existent, à titre expérimental s'il le faut, pour que nos habitants bénéficient d'un réel accès aux soins les plus vitaux à proximité de leur domicile. Concernant les difficultés de recrutement des médecins, puisque le salaire des médecins intérimaires doit être plafonné, le salaire des nouveaux médecins concourant à la permanence des soins dans ces structures pourrait bénéficier d'une surprime permanente en cas de travail de nuit. On peut également envisager l'ouverture de maisons médicales de garde sans condition d'un nombre moyen de passages aux urgences, ou encore l'aménagement du temps partagé de médecins salariés dans des centres de santé à l'hôpital. En outre, on

pouvez-vous me confirmer que l'hôpital de Sisteron et les autres hôpitaux du département auront bien des urgences de nuit ? Allez-vous soutenir la mise en place d'un nouveau modèle pour les urgences hospitalières de nuit dans nos territoires ruraux, fondé sur la proximité et adapté aux réalités géographiques et humaines de notre pays ? La parole

est confronté à des difficultés de recrutement dans un contexte national et départemental de raréfaction des ressources médicales, notamment urgentistes. Seul le service d'accueil des urgences est fermé la nuit. Le SMUR de l'établissement ainsi que l'unité d'hospitalisation La prise en charge urgente des patients sur le territoire est assurée. Le Chicas, dont dépend l'établissement de Sisteron, prévoit la mutualisation des postes d'urgentistes entre sites : une clause obligatoire a été ajoutée dans les contrats de recrutement des nouveaux praticiens intégrant l'établissement. Environ 20 % du temps de travail des urgentistes venant travailler à Gap devra être effectué sur le site de Sisteron. Par ailleurs, un projet de mutualisation des centres d'appel 15, du SAMU 04 et du SAMU 05 a vocation à apporter une réponse rapide à ce manque de ressources médicales.

Par ailleurs, le service d'accès aux soins déployé dès l'été 2020 doit garantir une réponse médicale de qualité en tous points du territoire.

Dans l'attente de cette réforme globale, vous avez annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros, qui permettrait aux conseils départementaux volontaires de commencer à mettre en oeuvre cette modulation positive à titre expérimental. Le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 est venu fixer le cadre de cette démarche.

le cadre du pacte de Cahors- et c'est bien là ma question -, a indiqué qu'il n'était « pas prévu de retraiter les dépenses exposées par les départements dans le cadre de la réforme de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ne correspondent ni à un transfert de compétences ni à un élément exceptionnel ».

L'aide à domicile constitue l'un des piliers de la réforme Grand âge et autonomie à venir. Elle vise à répondre à la préférence exprimée par nos concitoyens de pouvoir continuer à vivre chez eux.

Nous avons souhaité que, dès 2019, une enveloppe de 50 millions d'euros soit allouée aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, afin de préfigurer la mise en place d'un nouveau modèle de financement visant à améliorer la qualité du soutien à domicile, tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels. Cette enveloppe a été versée aux départements volontaires qui, comme vous le savez, sont chefs de file des politiques sociales, et dont nous voulons faire des acteurs de premier plan du maintien à domicile. Agnès Buzyn a récemment eu l'occasion d'évoquer ce sujet devant eux lors d'un séminaire organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le département du Loiret s'est engagé dans cette voie de l'amélioration des services à domicile, initiative qu'il faut saluer. Je précise que ces crédits, qui financent des dépenses de fonctionnement, relèvent bien du plafond défini par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. construire un partenariat renouvelé et renforcé avec les conseils départementaux. La réforme à venir pour le grand âge et l'autonomie doit nous permettre de renforcer les coopérations dans les territoires, pour garantir la qualité de l'accompagnement de nos aînés et de leurs aidants. La parole

aussi sur celle des médecins qui peuvent être les auteurs de tels accidents au cours de vies professionnelles, par ailleurs, parfaitement honorables. Ma question porte sur l'extension du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, et aux accidents médicaux faisant l'objet d'une réclamation au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, afin que celui-ci

Nous sommes sensibles à la situation de ces médecins et de leurs familles. Néanmoins, une extension de la garantie du fonds ne peut se faire que sous deux conditions : le respect absolu de l'indemnisation des patients et le maintien de l'équilibre financier du fonds. L'assurance fournie à certains praticiens pour des litiges passés ne doit pas nous pousser à prendre le moindre risque pour la viabilité de l'assurance future de leurs confrères et des victimes.

Elle porte sur la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouve le centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen depuis 2018. Ce centre hospitalier vit effectivement une période de crise durable qui ne cesse de s'aggraver à tous les points de vue. Tout d'abord, les locaux ne permettent plus d'assurer un accueil digne des personnes. L'occupation des lits dépasse largement la capacité de l'établissement. Ainsi, certains patients se retrouvent à dormir dans la salle de visite des familles ou dans des bureaux ; d'autres sont obligés de cohabiter dans des chambres très exiguës, le nombre de patients étant parfois trois fois plus élevé que l'unité prévue. Parallèlement, les conditions matérielles d'habitation sont déplorables : absence systématique de lunettes sur les cuvettes des toilettes, pas de sanitaires individuels. Les patients n'ont pas d'intimité : absence de serrure aux portes des chambres, portes avec des fenêtres de fermeture des placards. Par ailleurs, la liberté fondamentale d'aller et venir des patients est bafouée. La libre circulation des patients en soins libres dépend de la disponibilité des soignants : ils sont donc très souvent soumis à un enfermement injustifiable. Les patients en soins sans consentement sont privés de leurs droits, bien que les textes prévoient que toute restriction individuelle doit être décidée en fonction de l'état clinique du patient, après évaluation médicale. En outre, les pratiques d'isolement sont complètement illégales. L'isolement doit être une procédure de dernier recours. Or, dans de nombreux cas, la contention est la règle, et la liberté l'exception. Les conditions de rétention de ces patients sont particulièrement avilissantes : sans accès aux sanitaires, vous imaginez comment les choses se passent ! Sans accès aux personnels soignants, ils sont condamnés à se blesser physiquement en frappant à la porte autant de temps que nécessaire. patients sont également dessaisis de leur statut d'hospitalisation et de leurs droits. Ils ne disposent d'aucune information de la part des soignants sur l'offre de soins et les conditions de vie pendant leur séjour.

Comme vous le savez, le protocole d'accord signé entre la direction et les syndicats en juin 2018 prévoyait la création en priorité de trente nouveaux postes de soignants, dont le déploiement était prévu sur une année. La création de ces postes a fait l'objet d'un accord de financement intégral avec l'ARS Normandie pour un montant de 1,35 million d'euros. Conformément au protocole, les crédits correspondant aux vingt premiers postes ont été délégués et les recrutements intégralement effectués entre juin 2018 et juin 2019. L'ARS a délégué les crédits relatifs aux dix derniers postes en octobre 2019. Les professionnels concernés sont en cours de recrutement. Au-delà de ces moyens supplémentaires, le protocole prévoyait également la mobilisation des équipes médicale et soignante pour formaliser des projets en vue de l'amélioration des prises en charge.

par l'ARS. Il faut également accélérer le déploiement de nouveaux dispositifs de réhabilitation psychosociale selon un calendrier à définir. Enfin, il faut une actualisation du projet médical : l'établissement engagera dès le mois de janvier une révision de son projet médical l'appui d'un conseil extérieur, dans l'objectif de limiter strictement les restrictions à la libre circulation des patients à la mise en oeuvre du traitement requis. Soyez assurée, madame la sénatrice, que le

auteure de la question Dans un contexte de désertification médicale grandissante, nombreux sont les hôpitaux de proximité qui proposent des consultations réalisées par les praticiens exerçant au sein de ces établissements, ou bien par des médecins retraités qui acceptent de redevenir salariés des hôpitaux. Ils assurent ainsi l'offre de soins dans des secteurs en grande carence. Certes, l'activité externe n'est pas le coeur de métier de l'hôpital public, mais, si l'on s'en tient à la conception de l'hôpital de proximité telle que la développe votre gouvernement, ces établissements ont plus que jamais vocation à combler les manques existants, tout en favorisant bien sûr un partenariat et une dynamique avec les médecins libéraux locaux.

Les tarifs de ces actes et consultations externes à l'hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l'assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. Pourtant, à ce jour, les majorations tarifaires issues de ces conventions ne sont pas appliquées aux établissements de santé. En effet, un dispositif réglementaire limite nominativement les majorations transposables à l'activité d'actes et consultations externes des établissements de santé. Cette discrimination de traitement entre la ville et l'hôpital pour des soins pourtant similaires est injuste et préjudiciable, non seulement aux populations locales déjà dépourvues de médecins libéraux, mais également au budget de ces établissements de santé, souvent de petits hôpitaux en grande difficulté financière du fait de la tarification à l'activité (T2A) toujours pratiquée à ce jour. Cette discrimination entraîne la remise en cause de ces activités par ces petits hôpitaux largement sous-rémunérés selon l'inspection générale des affaires sociales. À l'heure où le financement au parcours est un élément constitutif de la stratégie nationale de santé, madame la secrétaire d'État, pensez-vous accorder aux établissements de santé un financement équitable de leurs actes et consultations externes, de manière à permettre cet ultime recours aux populations souvent rurales,

ce sur tous les territoires. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité, dans la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé votée l'été dernier, confier obligatoirement aux hôpitaux de proximité la mission de proposer des consultations de spécialités. Ces consultations pourront être assurées par des praticiens hospitaliers d'autres établissements dans le cadre de consultations avancées, ou par des praticiens libéraux du territoire des coopérations avec les cabinets de ville. Celles-ci pourront également être réalisées par télémédecine, notamment dans les territoires isolés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a permis de poser un modèle de financement adapté aux missions de ces hôpitaux, qui rompt avec la logique de la T2A. En effet, le financement de leur activité de médecine fera désormais l'objet d'une garantie pluriannuelle, qui assure à l'établissement de ne pas perdre de recettes sur la durée d'un cycle de trois ans, même si son activité venait à baisser. Ces hôpitaux bénéficieront aussi de crédits supplémentaires : la dotation de responsabilité territoriale d'exercer les missions d'appui au premier recours, de prévention, de prise en charge globale des personnes âgées qu'ils assurent en coopération avec l'ensemble des acteurs de leurs territoires. Vous avez raison de noter que l'offre de consultations externes, du fait de ses modalités techniques de financement, est parfois déficitaire pour des établissements de petite taille. Aussi l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 précise-t-il explicitement que cette dotation de responsabilité territoriale vise à soutenir l'offre de consultations de spécialités. Enfin, vous soulignez à juste titre l'asymétrie qui prévaut actuellement entre la ville et l'hôpital concernant l'application des majorations des conventions médicales. Ces dernières ne s'appliquent en effet aux établissements de santé que dès lors qu'elles ont été expressément prévues par un arrêté. À la suite de la publication de la convention médicale du mois d'août 2016, une réflexion sur l'ouverture progressive aux établissements de santé de l'ensemble des majorations tarifaires applicables aux actes et consultations externes a été lancée. Les travaux de transposition des majorations se poursuivent. Nous continuerons à mieux valoriser cette activité de

2019, le Gouvernement a présenté vingt-huit mesures pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, s'inspirant des conclusions du rapport présenté le 27 septembre 2018 par la mission d'information du Sénat sur les pénuries de médicaments et de vaccins, la situation ne s'améliore pas. Elle s'est même encore aggravée depuis la fin de l'été. Membre de cette mission d'information, je peux témoigner qu'un constat alarmant avait été dressé. Il y a plus d'un an, nous dénoncions déjà une mise en danger préoccupante de certains patients. sont à présent confrontés, tout comme les pharmaciens, à une grave pénurie de médicaments. Corticoïdes, antibiotiques, vaccins, la liste des médicaments en rupture de stock

Aujourd'hui, la rupture de stock du BCG-medac est effective. En France, les patients ne peuvent plus suivre leur traitement. Les urologues leur répondent qu'il faut patienter sans leur donner plus de précisions.

les signalements de tensions d'approvisionnement de médicaments ont été multipliés par vingt en dix ans. Face à ce constat et afin d'améliorer rapidement la situation, la ministre des solidarités et de la santé a présenté, le 8 juillet 2019, une feuille de route « lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France France », construite autour de quatre axes et de vingt-huit actions opérationnelles. Le comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments a été installé au mois de septembre. Il rassemble les associations de patients, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les médecins, les pharmaciens et les autorités nationales compétentes. Cette instance suivra l'évolution des travaux de la feuille de route menés dans le cadre des différents groupes de travail mis en place, et se réunira trois fois par an. En parallèle, compte tenu de l'impact des ruptures de stock dont vous avez rappelé l'effet pour certains médicaments, des mesures de prévention et de régulation ont été introduites à l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. D'une part, ces mesures visent à imposer, pour tout industriel, l'obligation de constituer un stock de sécurité qui ne peut excéder quatre mois pour tout médicament. D'autre part, le texte prévoit une obligation d'importation, aux frais de l'industriel, en cas de rupture d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave ou immédiat, ou en cas de rupture de stock d'un vaccin. J'ajoute que les sanctions concernant les manquements des industriels en cas de rupture de stock sont renforcées. Pour simplifier le parcours du patient, nous avons rendu possible le remplacement de médicaments par le pharmacien d'officine en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Par ailleurs, le Premier ministre a confié à M. Jacques Biot une mission visant à procéder à l'analyse des causes profondes de cette situation en matière de choix industriels. Il doit analyser les processus de production et

Madame la secrétaire d'État, j'entends bien votre réponse et vos arguments, mais je doute qu'ils satisfassent les patients, notamment ceux qui sont atteints d'une tumeur à la vessie.

de distribuer les unités par deux et non plus par six, la rupture de stock au 7 janvier 2020 est effective. Elle perdure depuis le 2 décembre 2019 et la remise à disposition n'interviendrait

Les 33 % d'honoraires de dispensation ne seront donc pas payés par les mutuelles, mais ils seront acquittés par les malades. Comme la prise en charge de la mutuelle n'est déclenchée qu'en cas de demande de remboursement à la sécurité sociale,

de l'honoraire du pharmacien, lequel ne sera pas pris en compte ? Sans compter que les sur-honoraires pour les médicaments prescrits aux enfants et aux personnes âgées sont passés à 3,5 euros et à 1,55 euro pour les anxiolytiques. an, je demandais déjà si l'information des patients sur cette situation pour le moins compliquée était prévue. Depuis un an, je suis allée un certain nombre de fois chez le pharmacien : je n'ai jamais

est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, permettez-moi tout d'abord de rappeler brièvement le contexte de mise en place de ces nouveaux honoraires. Une réforme du mode de rémunération des pharmaciens a été engagée avec la mise en place, en 2015, d'un honoraire au conditionnement et d'un honoraire pour pour ordonnance dite « complexe », facturé dès lors que les pharmaciens exécutent une prescription comportant au moins cinq lignes de médicaments différents remboursables, facturés à l'assurance maladie. Une seconde étape a été engagée avec l'avenant n° 11 en 2017, qui prévoit la mise en place de trois nouveaux honoraires de dispensation en en plus de ceux qui sont en vigueur depuis le 1 janvier 2015. S'agissant des conditions de prise en charge de ces honoraires par l'assurance maladie obligatoire, elles diffèrent selon le type d'honoraire. Pour l'honoraire au conditionnement, le taux de prise en charge est le même que celui du médicament dispensé, lequel dépend du niveau de service médical rendu (SMR). Pour les Pour les médicaments à SMR important, le taux est fixé à 65 % ; pour ceux à SMR modéré, le taux est de 30 % ; pour ceux à SMR faible, le taux est de 15 %. Pour l'honoraire pour ordonnance dite « complexe », la participation de l'assuré est supprimée. Pour les trois nouveaux honoraires de dispensation, le taux de prise en charge par l'assurance maladie est de 70 %, soit une participation de l'assuré de 30 %. Pour ce qui concerne les modalités d'information sur les prix des médicaments et les honoraires de dispensation dans les officines de pharmacie, elles sont fixées par un arrêté du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, datant du 28 novembre 2014 et publié le 4 février 2015. Ce texte sera mis à jour en 2020 pour, notamment, intégrer les nouveaux honoraires de dispensation mis en place depuis le 1 janvier 2019. Enfin, la liste des médicaments dit « spécifiques » faisant l'objet d'un honoraire de dispensation particulière figure en annexe II.4 de l'avenant n° 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie.

Madame la secrétaire d'État, la grande majorité des associations représentatives des personnes handicapées est très défavorable à l'intégration de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le revenu universel d'activité (RUA) annoncée par le Gouvernement. Ces associations estiment à bon droit que l'AAH est non pas un minimum social, mais une prestation sociale liée à la reconnaissance d'une incapacité spécifique souvent, hélas, pérenne. Intégrer l'AAH dans le RUA serait non seulement une remise en cause fondamentale des droits des handicapés et du cadre législatif acté en 1975 et en 2005, mais entraînerait de surcroît très vraisemblablement une dégradation des droits des bénéficiaires de cette prestation, alors alors même que, dans le cas d'une politique réellement inclusive, le montant actuel de l'AAH mériterait grandement d'être réévalué au regard des besoins des personnes handicapées. Entendez-vous prendre en compte ces inquiétudes et renoncer à l'intégration de l'AAH dans le RUA ? dans le RUA ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question importante du revenu universel d'activité et de l'inscription de l'allocation aux adultes handicapés au sein des concertations ouvertes ouvertes en juin dernier sur le revenu universel d'activité. Ce minimum social, témoin de la solidarité nationale, a été très fortement revalorisé par le Gouvernement. Comme vous le savez, la hausse s'élève à plus de 11 %.

Cette réforme fait l'objet d'une concertation institutionnelle et citoyenne afin de permettre une large consultation de l'ensemble des personnes intéressées. La concertation institutionnelle s'appuie sur différents collèges. Le 4 juillet dernier, Sophie Cluzel a lancé les travaux du collège thématique dédié aux personnes en situation de handicap. Ce n'est qu'à l'issue de cette concertation que le périmètre de la réforme sera arrêté. Aucune décision n'est donc prise concernant l'AAH. L'objectif du revenu universel d'activité étant de lutter contre la pauvreté et de la faire reculer, le Gouvernement ne portera en conséquence aucune réforme qui pénaliserait les plus vulnérables. Cependant, exclure de cette réflexion transversale à l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux le champ du handicap fermerait le dialogue sur les questions de la pauvreté et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, privant notamment les jeunes d'un l'activité. Je rappelle que le revenu universel d'activité vise deux objectifs très clairs : l'accompagnement vers l'activité et l'assurance qu'une reprise d'activité se traduira par un gain.

notamment dans le cadre des concertations. Les allocataires de l'AAH ne s'inscrivent pas dans une conditionnalité de reprise d'activité. Le bénéfice du revenu universel d'activité ne sera donc pas attaché à une obligation de recherche et de reprise d'activité pour les personnes en situation de handicap.

et pour chacun les mesures adaptées pour tendre vers l'équité. Telle n'est pas, à l'évidence, la philosophie du RUA. On verra d'ailleurs bien ce qu'il en adviendra. Quoi qu'il en soit, je vous en conjure : l'AAH ne peut pas et ne doit pas disparaître au profit du RUA, car-

Il s'inscrit dans le préambule de notre Constitution, qui dispose que « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Ainsi, sur les 1 849 volontaires retenus pour expérimenter ce nouveau dispositif, plus de 850 personnes durablement privées d'emploi ont été embauchées dans le cadre d'un contrat de travail classique ou ont retrouvé un emploi. Plus de 20 % d'entre elles avaient un handicap qui rendait leur insertion professionnelle encore plus difficile. De plus, cette expérimentation a un effet d'émulation sur chacun des territoires concernés, comme j'ai pu le constater à Mauléon, dans mon département des Deux-Sèvres. Madame la secrétaire d'État, je suis étonné que le projet de loi d'extension de ce dispositif ne soit toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Le Président de la République avait annoncé en septembre 2018, lors de la présentation de la stratégie de lutte contre la pauvreté, l'extension de l'expérimentation à 50 nouveaux territoires. Il a également insisté le 1 mars 2019, à Bordeaux, lors d'un grand débat, sur l'urgence d'étendre le dispositif. Plus d'une centaine de territoires se sont déjà déclarés volontaires et sont dans l'attente de l'adoption de ce texte. Par ailleurs, 200 parlementaires soutiennent cette initiative et la Belgique s'apprête à expérimenter le projet. social et environnemental) d'une demande d'avis sur la prévention et la réduction du chômage de longue durée, faisant référence à cette expérience. L'extension du dispositif restait suspendue aux conclusions de rapports qui, aujourd'hui, sont connues.

S'agissant de l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée prévue par la loi du 29 février 2016, elle a été lancée de manière opérationnelle en janvier 2017. Nous en sommes donc à trois années tout juste de mise en oeuvre. Depuis 2017, douze entreprises à but d'emploi (EBE) ont été créées sur les dix territoires qui ont été retenus après appel à projets. Ce sont 900 personnes privées d'emploi qui ont pu être recrutées, dont 750 sont actuellement salariées.

seront financés en 2020, en cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. La contribution totale de l'État s'élève à 28,5 millions d'euros dans le cadre de la loi

Comme toute expérimentation, il est désormais important de prendre du recul pour l'évaluer et partager avec tous les acteurs un diagnostic. C'est dans ce sens que Muriel Pénicaud a réuni lundi 25 novembre dernier

pour une grande part, qu'il s'agisse des fragilités comme des points positifs. C'est pourquoi Muriel Pénicaud a demandé à l'association qui porte l'expérimentation et à ses services de poursuivre le travail de diagnostic- une réunion a eu lieu en décembre -pour permettre, dans les prochaines semaines, de faire des annonces sur les suites à donner à cette expérimentation. La parole

La commune de Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime, et son agglomération Caux Seine Agglo ont développé une méthodologie tendant à mettre en place cette expérimentation sur un territoire extrêmement dynamique. L'engagement des collectivités locales est fort pour trouver des solutions innovantes en parallèle des actions de développement économique et d'attractivité du territoire de la vallée de la Seine.

Les résultats sont encourageants. Le taux de chômage, certes encore très élevé dans notre pays, a baissé de 9,6 % à 8,6 %, soit son plus bas niveau depuis dix ans. Le nombre de créations d'emplois nettes s'élève à 258 cette année et à 540 000 depuis deux ans et demi. S'agissant de l'apprentissage, les résultats sont historiques : 458 000 apprentis, soit 8,4 % de plus au premier semestre 2019. Ces résultats nous invitent à poursuivre l'effort, notamment à l'égard des jeunes, sujet que vous suivez attentivement au

visant à résorber le chômage de longue durée. Ainsi, 1 000 équivalents temps plein supplémentaires seront financés en 2020, en cohérence avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La contribution totale de l'État s'élève à 28,5 millions d'euros, soit 6,13 millions d'euros de plus

Les auto-écoles dites « traditionnelles » subissent la concurrence de nouveaux prestataires sur internet, qui proposent des prix paraissant plus attractifs. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes charges qui pèsent sur les uns et sur les autres. Les auto-écoles telles que nous les connaissons assurent un emploi stable à leurs personnels, paient des charges sociales, les véhicules, le carburant et les assurances. Sur internet, les prestataires mettent en relation les élèves avec un moniteur auto-entrepreneur ou indépendant qui exerce à son compte. Avec ce mode de fonctionnement, l'État perd des ressources fiscales et sociales ; pour les personnels, les emplois deviennent précaires. Si, par exemple, les auto-écoles traditionnelles venaient à disparaître dans mon département de l'Aveyron, de l'Aveyron, il n'est pas sûr que des auto-entrepreneurs viennent proposer des heures de conduite. Pour passer le permis de conduire, les élèves devraient effectuer de nombreux kilomètres avant de pouvoir trouver un de ces nouveaux moniteurs.

Comme vous le savez, le secteur de l'éducation routière a été profondément bouleversé ces dernières années. L'émergence des nouveaux modèles en ligne, à condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la loi et d'un apprentissage de qualité, peut constituer un complément à l'offre proposée dans nos territoires. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause le modèle auquel nous sommes attachés et qui favorise le lien social. Les réformes entreprises depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont permis de nombreuses avancées. Je pense, par exemple, à la réduction significative des délais de passage aux examens. À cet égard, je tiens à saluer l'engagement de nos 1 400 inspecteurs du permis et leur capacité à s'adapter en permanence aux nouveaux défis. Dans la continuité des travaux engagés, un plan de réforme constitué de dix mesures, vous l'avez rappelé, a été présenté le 2 mai 2019 par le Premier ministre. Sur ces dix mesures, trois sont déjà entrées en vigueur : le développement de l'usage du simulateur de conduite dans la formation, qui requiert un local, le développement de l'apprentissage de la conduite sur boîte automatique et l'abaissement de l'âge de passage de l'examen dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. Les sept autres mesures sont en cours de déploiement. Portées notamment par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, elles concernent la gratuité de l'examen théorique pour les volontaires du service national universel, la mise en place place d'une plateforme gouvernementale dédiée au choix de son auto-école, le développement des apprentissages accompagnés de la conduite, la mise en place d'une nouvelle épreuve théorique moto du code de la route, la modernisation de l'inscription à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire ou encore la mise en place d'un livret d'apprentissage numérique. Vous le constatez, le Gouvernement poursuit sa politique innovante et veille à ce que, quel que soit le modèle économique choisi, soient garantis un enseignement de qualité et la sécurité des apprentis conducteurs. La parole

ont été touchées par des mouvements de terrain, ce qui provoque de véritables drames humains. Confronté à un risque d'effondrement, le maire de Leforest n'a eu d'autre choix, sa responsabilité étant engagée, que de prendre un arrêté de péril imminent, synonyme, pour d'expulsion, donc de désarroi moral et matériel, les intéressés devant continuer à rembourser leur crédit immobilier. Jusqu'en décembre dernier, leur seul espoir était que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour 2018, afin que les assurances puissent les indemniser.

vous avez appelé mon attention sur la situation de la commune de Leforest, dans le Pas-de-Calais, qui a déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2018. Par arrêté interministériel du 15 octobre 2019, publié au le 15 novembre 2019, Je souhaite vous préciser que, pour décider de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour une commune, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts, et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes. Ces critères techniques sont fondés sur des études approfondies réalisées par les services d'expertise mandatés par l'administration. Chaque commune touchée par le phénomène et ayant déposé une demande fait l'objet d'un examen particulier. Compte tenu de la cinétique lente qui caractérise l'aléa de sécheresse et des connaissances scientifiques disponibles à ce jour, il est considéré que ces phénomènes, engendrés par le retrait et le gonflement des argiles, ne peuvent se produire que si deux conditions se trouvent conjointement remplies d'une part, une condition géotechnique- un sol d'assise des constructions constitué d'argiles sensibles au phénomène de retrait et de gonflement -, et, d'autre part, une condition de nature météorologique, à savoir une sécheresse du sol d'intensité anormale. La méthode appliquée pour instruire les demandes communales formulées au titre de ce phénomène a été révisée par une circulaire datée du 10 mai 2019 afin, d'une part, de tenir compte des progrès les plus récents dans la modélisation hydrométéorologique réalisée par Météo France, et, d'autre part, de fixer des critères plus plus lisibles, pour les municipalités et pour les sinistrés, de caractérisation de l'intensité d'un épisode de sécheresse et réhydratation des sols. Cette nouvelle méthode a été mise en application pour traiter l'ensemble des demandes communales déposées au titre de l'épisode de sécheresse de 2018.

En revanche, au regard des données recueillies par Météo France, les niveaux d'humidité des sols superficiels de Leforest ne relèvent d'une sécheresse géotechnique anormale pour aucune des quatre saisons de l'année 2018. Je ne méconnais pas les effets des mouvements différentiels de terrain provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols sur certains immeubles de Leforest, mais seuls les épisodes de sécheresse présentant une intensité anormale avérée donnent lieu à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui n'est malheureusement pas le cas de cette commune pour l'ensemble de l'année 2018. La parole

je vis en Meurthe-et-Moselle, à Villerupt, une commune d'environ 10 000 habitants située à une trentaine de kilomètres, par la route, de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, et à 5 kilomètres de la ville d'Esch-sur-Alzette, au Luxembourg.

toute la population est progressivement dotée de pastilles d'iode en prévision d'un éventuel accident à Cattenom : un comble quand on sait que les habitants du Luxembourg sont plus éloignés de la centrale que ceux de ma commune et de nombreuses autres communes de mon département ! Comme je le disais, la règle retenue, qui repose sur le seul kilométrage,

éventuellement exposées. Si la prise de pastilles d'iode ne permet pas, on le sait, de parer à un accident, elle constitue une solution d'urgence permettant d'éviter en partie le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive.

depuis 1997, des campagnes de distribution de comprimés d'iode aux riverains des centrales nucléaires sont régulièrement organisées. Elles concernent effectivement les zones situées dans un rayon de 10 kilomètres autour d'une centrale et intégrées au plan particulier d'intervention (PPI).

Dans le cadre de l'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) aux échelons zonal et départemental, cette prédistribution est complétée par le prépositionnement de 110 millions de comprimés. Le prépositionnement, instauré dans les zones où l'urgence est moindre, offre une meilleure traçabilité et de meilleures conditions de stockage ; il permet surtout de déplacer rapidement les stocks, lesquels sont suffisants pour couvrir l'ensemble de la population. Ce sont les préfets qui organisent les plans de distribution des comprimés. S'ils estiment que la situation nécessite la prise de comprimés, les stocks sont déployés vers des points de distribution. Les campagnes de distribution de comprimés d'iode permettent de sensibiliser aux risques et de mobiliser les citoyens, dont l'implication est indissociable d'une gestion efficace des crises. De nombreux acteurs de

et les carences sont bien réelles. La banque publique de la démocratie doit devenir une réalité, utile non aux seuls partis, mais bien à notre démocratie. Les pistes sont nombreuses

a pour mission de contribuer à rapprocher les candidats, partis et groupements politiques et les banques. Dans son rapport rendu le 30 septembre dernier, à la suite des élections européennes du 26 mai 2019, le médiateur n'a pas relevé de difficultés systémiques, corroborant ainsi l'analyse menée en 2017 ce rapport a mis en lumière que, sur les trente-quatre listes de candidats aux élections européennes, huit ont été confrontées à des difficultés pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, alors même que le législateur garantit un droit au compte, tandis que neuf partis ont essuyé un refus de prêt bancaire. Ces chiffres révèlent une situation perfectible et le médiateur a fait plusieurs propositions de nature à la faire évoluer. Il appelle notamment à la réduction des délais pour les ouvertures de comptes bancaires, pour la délivrance des moyens de paiement et pour l'instruction des demandes de prêt. il est important que les candidats et les partis connaissent mieux les critères et exigences des établissements bancaires. Le site internet de la médiation, en cours de construction, devrait faciliter l'information sur les dispositifs en vigueur ou en cours de mise en place. Au-delà de ces actions de sensibilisation, le médiateur a fait plusieurs recommandations visant à élargir l'accès de tous les candidats à la propagande, ce qui passe notamment par un surcroît de dématérialisation. Par ailleurs, le rapport du 30 septembre 2019 met l'accent sur la nécessité, pour les candidats et les partis politiques, de recourir aux autres modalités de financement qui leur sont ouvertes, au-delà des aides publiques : appels aux dons de sympathisants et militants, emprunts auprès des partis et, désormais, auprès des particuliers. Cette dernière modalité a d'ailleurs été largement mise en oeuvre lors des récentes élections européennes. De même, en application de la loi du 2 décembre dernier, qui entrera en vigueur le 30 juin 2020, les partis et candidats pourront recueillir des fonds un financement participatif.

à M. le ministre de l'intérieur. Conformément à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie, un règlement départemental a été approuvé par la préfecture de Seine-Maritime

y compris en optant pour des bâches extérieures, pourtant moins coûteuses. Le référentiel national ne tient pas compte des spécificités locales, ce qui complexifie encore la situation. Il interdit par exemple le recours aux dispositifs mobiles des sapeurs-pompiers, qui serait pourtant particulièrement adapté pour les habitations isolées. Encore une fois, les élus locaux ont l'impression que les décisions prises sont déconnectées de la réalité des territoires ; c'est pourquoi ils avaient rejeté, en 2017, une première proposition de règlement départemental. L'application stricte des distances retenues rend la situation intenable en Seine-Maritime. Pour beaucoup de maires, cela implique de cesser d'accorder des permis de construire et même, souvent, de se retrouver

en eau et les ressources disponibles. La défense extérieure contre l'incendie (DECI), placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à couvrir, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Il s'agit d'un appui indispensable pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement, efficacement et dans des conditions optimales de sécurité. La réforme de la DECI, conduite en 2015, a instauré une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif : un renforcement de la concertation avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et l'application des mesures, adaptées à la réalité et à la diversité des risques incendie propres à chaque territoire. La distance maximale séparant les points d'eau et les risques à couvrir est déterminée au regard des enjeux en matière de protection et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers. La fixation de ces distances est déterminée par l'analyse du risque d'incendie et elle conditionne les délais de mise en oeuvre des dispositifs d'extinction. J'ai parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes, notamment rurales. Ce règlement peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables. J'ajoute que la DECI ne doit pas altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée ni conduire à des dépenses excessives, au regard, notamment, du dimensionnement des canalisations. Si le réseau d'eau potable ne permet pas d'obtenir le débit nécessaire à la DECI, d'autres ressources sont utilisables : points d'eau naturels, réseaux d'irrigation agricole, citernes fixes, cuves ou encore réservoirs réalimentés par l'eau de pluie. La DECI repose sur un équilibre entre les impératifs de la sécurité des populations, sa constante amélioration et un coût financier supportable, notamment pour les communes rurales, le tout étant apprécié à l'échelon local. La parole

que je représente ici, sur la reconnaissance du tilde dans les actes de l'état civil et sur la date prévisible de l'ajout de ce signe à la liste des signes diacritiques admis en langue française au travers de la circulaire du 23 juillet 2014. Tout d'abord, il faut souligner que la promotion des langues régionales est assurée de diverses manières et, ainsi que le rappelle notamment le contrat d'action publique pour la Bretagne, elle passe principalement par le biais de l'enseignement et de la culture. La circulaire du 23 juillet 2014 de la Chancellerie que vous évoquez dresse la liste des voyelles et consonne accompagnées d'un signe diacritique souscrit- placé au-dessous de la lettre, telle la cédille -ou suscrit- placé au-dessus de la lettre, tels l'accent et le tréma -connues de la langue française. Cette liste, ne comprenant pas le tilde, a été validée en 2014 par l'Académie française, qui a confirmé sa position en novembre 2018. Le 17 octobre 2019, dans l'affaire Fañch, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, au motif que les parents de l'enfant n'avaient été appelés qu'en leur qualité personnelle, et non en leur qualité d'administrateurs légaux de l'enfant. Ainsi, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire ni sur la possibilité d'employer le tilde dans les actes de l'état civil, en l'occurrence sur la lettre « Néanmoins, nous souhaitons indiquer que, pour ce qui concerne l'état civil, les services de l'État étudient la faisabilité d'une intégration de signes diacritiques pour permettre la prise en compte de l'orthographe de certains prénoms issus de langues régionales au regard, d'une part, des enjeux normatifs et informatiques, et, d'autre part, de la charge de travail des officiers de l'état civil. Enfin, dans la continuité des actions de promotion des langues régionales de France, les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, autorisent les officiers de l'état civil à délivrer, sur la demande des intéressés, des livrets de famille et des copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil bilingues

sont de plus en plus fréquentes. Ces violences sont inacceptables. Entre 2017 et 2018, plus d'une centaine d'actions illégales ont eu lieu partout en France. Bien évidemment, je respecte les idées de ces militants, mais eux doivent respecter nos agriculteurs, dont les activités sont, elles, légales. Dans leur immense majorité, nos agriculteurs veillent au bien-être animal.

Une prise de conscience et une mobilisation collectives des professionnels et des élus sont indispensables pour dénoncer ces agissements. Dans mon département, la Mayenne, un observatoire de l'agri-bashing a été mis en place. Il rassemble les services de l'État, les syndicats agricoles et la chambre d'agriculture en vue de lutter contre les intrusions dans les exploitations. Les filières agricoles et agroalimentaires attendent des réponses très concrètes de la part de l'État : une évolution de la loi doit permettre de prononcer des sanctions fermes contre les malfaiteurs qui, par leurs intrusions dans les exploitations, bafouent la propriété privée.

qui concerne tout notre territoire. Le Gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre les actions violentes que subissent certains professionnels de la filière agroalimentaire. À ce titre, la direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé, le 22 février 2019, une dépêche sur le phénomène des actions violentes de mouvements animalistes radicaux, afin de mobiliser les parquets et de leur rappeler les qualifications pénales pouvant être retenues dans ces situations. Ces agissements font ainsi l'objet de la plus grande attention de la part des procureurs, qui diligentent systématiquement des enquêtes pénales minutieuses, aux fins d'établir le contexte de la commission des faits, d'en identifier les auteurs et de présenter ces derniers à une juridiction.

similaires à ceux que vous évoquez, qui ont pu avoir lieu ailleurs sur notre territoire national, ont d'ailleurs déjà conduit à des condamnations. Par exemple, en décembre 2018, six personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Roanne du chef de violation de domicile alors qu'elles avaient pénétré sur un site d'abattage sans autorisation ; en juin 2019, le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux individus à trois mois et six mois d'emprisonnement pour des dégradations commises dans une boucherie parisienne et des violences sur les personnes d'un boucher et de fromagers. Ces réponses judiciaires attestent de la prise en compte par les parquets du trouble à l'ordre public inacceptable ou de l'entrave à l'exercice professionnel qu'occasionnent de tels agissements, nécessitant, lorsque les éléments de preuve recueillis le permettent, une réponse pénale ferme et adaptée. Le ministère de la justice estime que le cadre juridique actuel permet, dans la plupart des cas, de répondre efficacement aux actions violentes subies par les professionnels de la filière animale.

du délit de violation de domicile pour lever toute ambiguïté sur le fait que ce délit trouve bien à s'appliquer, y compris en cas d'intrusion dans les locaux professionnels d'une exploitation agricole. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour la réplique.

Selon les enquêteurs, le véhicule des ravisseurs serait tombé en panne et ces quatre hommes auraient éliminé les deux otages avant de prendre la fuite. Plusieurs zones d'ombre demeurent dans cette affaire tragique.

ce qui pourrait laisser penser qu'il aurait été recruté comme informateur par les services de la DGSE. Qu'en est-il, monsieur le secrétaire d'État ? Deuxièmement, différentes enquêtes effectuées par les journalistes mettent en avant un lien possible, et même probable, entre cet assassinat et l'affaire Arlit, désignant l'enlèvement d'employés d'Areva en 2010 au Niger. Selon ces enquêtes, leur libération aurait été négociée en échange d'une rançon de 30 millions d'euros et l'enlèvement des deux journalistes aurait été commis par des membres d'un bataillon considérant avoir été floués dans la répartition de cette rançon. Qu'en est-il ? Troisièmement, il existe deux versions contradictoires sur un fait essentiel : les autorités françaises ont formellement assuré que les militaires étaient arrivés sur place n'avaient jamais eu de contact avec les ravisseurs ; un rapport des Nations unies affirme strictement le contraire. Quelle est la vérité ?

ont indiqué être intervenus sur une scène de crime largement souillée et modifiée, alors que le détachement de Serval avait reçu l'ordre de ne toucher à rien. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet

Claude Verlon. Ces faits d'enlèvement et d'assassinat font l'objet d'une information judiciaire, dans le cadre de laquelle le ministère des armées a apporté et continue d'apporter son plein concours. Les forces françaises ont toujours appuyé l'action judiciaire, que ce soit sur place, à Kidal, au lendemain des faits, ou à Paris. Je rappelle que c'est avec le concours de l'armée française, dans un contexte sécuritaire tendu, que les gendarmes de la prévôté ont été projetés sur les lieux, pour effectuer les premières constatations et fournir à la justice le maximum d'éléments de preuve. Les enquêteurs français de la direction centrale du renseignement intérieur de l'époque et de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ont également pu intervenir très rapidement. Cet appui logistique assuré dès le départ s'est poursuivi à mesure des besoins exprimés par les magistrats. En effet, le ministère des armées a été requis à plusieurs reprises, en 2015 et en 2016, par les magistrats chargés de l'enquête. Toutes les demandes de déclassification successives formulées par la justice ont donné lieu à la fourniture de documents du ministère des armées, en parfaite conformité avec les avis de la Commission du secret de la défense nationale, qui est une autorité administrative indépendante. Si des documents ou extraits de documents n'ont pas été déclassifiés, c'est uniquement, comme le prévoit la loi, pour préserver les capacités et méthodes des services, mais aussi assurer la continuité des opérations ou la protection des personnels. Conscient de la douleur des proches des journalistes assassinés, le ministère des armées a, autant que le lui permet l'impératif de protection du secret de la défense nationale et de l'instruction, répondu directement aux interrogations de ces derniers. Je vous le redis, monsieur le sénateur, le ministère des armées continue à appuyer les investigations judiciaires en cours et répond avec une extrême diligence aux sollicitations des magistrats. En revanche, cet appui n'a pas vocation n'a pas vocation à être exposé publiquement, car il est couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction. Je pense que vous le comprendrez. La parole

décédée « du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». Cependant, l'appréciation des « circonstances exceptionnelles » est laissée au ministre en fonction. Or, avant 2017, les attributions de la mention « mort pour le service de la Nation » ont confirmé la reconnaissance des militaires décédés « accidentellement » lors d'exercices opérationnels. depuis cette date, les décisions de la ministre vont à l'encontre de l'esprit initial du décret du 28 décembre 2016. En effet, les demandes de mention « mort pour le service de la Nation » pour des militaires qui décèdent accidentellement lors d'exercices opérationnels ou en missions intérieures sont désormais systématiquement rejetées.

de ces derniers ne sont pas reconnus comme « pupilles de la Nation », leur conjoint ne perçoit que 50 % de la pension de réversion et leur nom ne sera pas gravé sur le monument aux morts de leur commune. L'un de mes collègues députés a déposé, le 22 mai dernier, une proposition de loi visant à octroyer le statut de « mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en exercice, ce qui permettrait d'assainir la situation actuelle et de la rendre plus juste.

pour le service de la Nation » afin de supprimer l'arbitraire et d'intégrer les militaires décédés accidentellement lors d'exercices opérationnels ou en missions intérieures. Cela permettrait d'assurer notre soutien fraternel aux familles de ceux qui s'engagent pour défendre notre pays.

d'attribution de la mention « mort pour le service de la Nation ». Cette mention a été créée en 2012, au lendemain des attentats commis par Mohammed Merah contre la communauté juive et contre l'armée. Elle vise à honorer la mémoire des militaires et des agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité par l'action volontaire d'un tiers. Vous avez évoqué le décret de 2016, qui est venu inclure le décès « dans des circonstances exceptionnelles », appréciées comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormale et imprévisibles. Les mesures symboliques prises par la République n'ont de valeur que si elles sont précisément ordonnées. Le décret de 2016 a créé des incertitudes, et le ministère des armées réfléchit à la façon dont il peut y mettre fin pour éviter toute confusion et tout sentiment d'injustice. il n'est pas souhaitable, pour la mémoire et la reconnaissance des militaires tués au combat ou celle des agents publics victimes d'actes de terrorisme, d'étendre de façon indéfinie l'attribution des marques de reconnaissance. Les armées sont légitimement attachées à ces distinctions et à leur sens. Toutes les morts sont tragiques. Le ministère des armées s'attache à apporter un soutien sans faille aux familles endeuillées. Les ayants cause peuvent ainsi se voir attribuer une allocation du fonds de prévoyance. Les enfants mineurs peuvent également bénéficier d'un régime de protection particulier.

et, à travers lui, le Gouvernement -apporte un soutien fraternel aux familles de tous les militaires décédés, que ce soit en combat ou en accident de service. Toutefois, il n'envisage pas d'étendre à ce dernier cas l'attribution de la mention « mort pour le service de la Nation ». La parole

Je prendrai l'exemple du flamand occidental, parlé dans mon territoire des Flandres françaises, mais je pense aussi au picard, cher à mon ami Jérôme Bignon, et à toutes les autres langues de France. Le Gouvernement tente de mettre en oeuvre, depuis 2017, le programme défendu par Emmanuel Macron lors de la campagne pour la dernière élection présidentielle et les engagements pris à cette occasion.

scolaire de ces langues régressent ... et la promesse du Président de la République est bafouée. Un exemple illustre le renoncement du Gouvernement à protéger les langues minoritaires. Dans les Hauts-de-France, le flamand occidental bénéficiait d'un enseignement depuis dix ans. Expérimenté pendant trois ans, celui-ci avait été validé après une évaluation rigoureuse. Suivi dans plusieurs écoles de l'arrondissement de Dunkerque, cet enseignement était très apprécié des jeunes et de leurs familles et complété par des activités extrascolaires, preuve de l'intérêt de la population. L'heure de la retraite est venue pour l'enseignant

C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à attendre votre réponse à la question suivante : que compte faire le Gouvernement pour encourager l'apprentissage des langues régionales sur les territoires qui ont la chance d'en posséder une ? Plus précisément, pour le cas du flamand occidental, entendez-vous remplacer

qui ne fait pas l'objet d'un enseignement de langue et culture régionales tel que décrit dans la circulaire du 12 avril 2017. Rappelons d'abord que l'introduction d'un nouvel enseignement de langue vivante dans notre système scolaire, de l'école primaire au baccalauréat, doit être étudiée au regard de nombreux critères, tels que sa zone d'implantation et de diffusion, le nombre de locuteurs potentiels et le degré d'imprégnation et d'utilisation de la langue par la population, le corpus disponible dans les différents registres littéraires ou encore la demande des familles. Ainsi, la situation du flamand occidental doit être appréciée avec finesse et discernement au regard de l'ensemble de ces éléments. En outre, vous le savez bien, monsieur le sénateur, l'enseignement du néerlandais, langue de communication avec la Région flamande de Belgique et les Pays-Bas, est une priorité de l'académie de Lille, notamment pour le département du Nord, aussi bien pour l'enseignement primaire que pour le collège et le lycée. L'apprentissage de cette langue répond notamment à de forts enjeux économiques et d'employabilité. De fait, c'est la connaissance de la langue néerlandaise qui permet aux élèves de la zone frontalière de trouver des débouchés professionnels, ce qui n'exclut pas, bien sûr, une connaissance de ses variations dialectales. La sensibilisation à la langue et à la culture du flamand occidental peut trouver une place à l'école. Le code de l'éducation dispose que les enseignants des premier et second degrés « sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. » Cette sensibilisation peut intervenir en classe, durant le temps scolaire, dans le cadre de plusieurs enseignements, notamment de langues vivantes, par exemple en cours de néerlandais, d'histoire, d'enseignement artistique ou d'histoire de l'art. Ainsi, la proximité linguistique de la langue régionale flamande avec la langue néerlandaise peut être avantageusement mise à profit lors des séances consacrées à l'apprentissage de cette dernière, avec un travail sur les nuances dialectales et sur les réalités culturelles de l'espace linguistique du franco-flamand. Les enseignements pratiques interdisciplinaires du collège, qui réunissent plusieurs disciplines autour de projets communs, souvent ancrés dans les réalités locales, offrent un cadre propice à une telle sensibilisation. Signalons aussi qu'un enseignement de la variante française du flamand occidental est dispensé dans trois écoles primaires publiques dans le cadre d'une expérimentation. La poursuite de cette expérience sera fonction des conclusions de l'évaluation qui sera conduite par les services de l'académie de Lille. Enfin, à l'école primaire, la sensibilisation au flamand occidental et à la culture qu'il porte peut aussi faire l'objet d'activités éducatives et culturelles complémentaires, conduites dans les temps périscolaires, en lien, par exemple, avec des associations locales bénéficiant d'un agrément pour intervenir en milieu scolaire. La parole

Il n'y a pas d'antagonisme entre le néerlandais et le flamand. Le flamand est d'ailleurs antérieur au néerlandais. Pourquoi réserverait-on un traitement particulier à cette langue régionale qu'est le flamand occidental ?

et de l'alimentation. Ma question porte sur le développement de l'agroforesterie. En Guadeloupe, la culture de la banane et celle de la canne à sucre sont fragilisées, depuis plusieurs années, par un contexte économique et social difficile, ainsi que par l'âpre concurrence des pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. Il convient, dans ce contexte, de repenser en partie le développement de notre filière agricole. Certaines cultures traditionnelles de niche- je pense notamment au café, au cacao et à la vanille -offrent, par exemple, des perspectives intéressantes. Principalement destinées à l'exportation, ces cultures de sous-bois, en nombre limité aujourd'hui, pourraient permettre à la Guadeloupe de diversifier sa production agricole sans rogner sur les cultures déjà existantes, et ce malgré la réduction du foncier disponible. L'agroforesterie est également pourvoyeuse d'emplois, puisque les exploitations, non mécanisées, doivent recourir à de nombreux salariés agricoles. Son développement permet, en outre, de répondre à certaines considérations environnementales. Un projet d'implantation d'un parc agroforestier et agrotouristique a ainsi vu le jour sur le territoire de Bouillante, en Guadeloupe. D'autres ne demandent qu'à émerger. Cependant, le fait que l'agroforesterie relève de la foresterie, et non pas de l'agriculture, freine son développement, en Guadeloupe comme ailleurs. Il en résulte une baisse importante des financements alloués à ces projets. Envisagez-vous, monsieur le ministre, de faire évoluer cette classification, afin de favoriser le développement de cette activité ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le

et de l'alimentation a diffusé une instruction rappelant notamment « la nécessité d'éviter la consommation de ces denrées par les jeunes enfants, particulièrement en restauration collective », « que les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer ces produits » et que « les qualités nutritionnelles de ce type de produits » ne peuvent « occulter le risque sanitaire ». Bien entendu, je ne remets pas en cause le bien-fondé de ces recommandations. Il est vrai qu'une trentaine de cas d'infections et un dramatique décès ont été portés à la connaissance des pouvoirs publics en mai 2018 2018 et en avril 2019. Il est évidemment responsable et attendu que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation prévienne ces risques et alerte à leur sujet. Néanmoins, vous devinez, monsieur le ministre, que cette application stricte du principe de précaution conduit une grande partie des responsables de restauration collective à ne prendre aucun risque et donc à ne plus offrir ces produits. Dans un contexte où la défiance envers les agriculteurs et les éleveurs est telle qu'ils dénoncent l'agri-bashing dont ils sont victimes, cette mesure distend un peu plus le lien entre société et agriculteurs. Pourtant, de nombreuses collectivités locales sont engagées avec les producteurs locaux dans une démarche de circuits courts et d'intégration de leurs produits dans la restauration collective. Ainsi, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, comme beaucoup d'autres, est le promoteur, auprès des communes et des intercommunalités, de la belle démarche « Manger bio & local, labels et terroirs ». L'éducation nationale, quant à elle, favorise l'éducation au goût. Les semaines du goût dans les établissements scolaires connaissent un grand succès. Il serait donc paradoxal que l'instruction de votre ministère freine le recours à la production locale et conforte la prééminence de la nourriture industrielle dans la restauration collective, laquelle n'est pas non plus imperméable aux difficultés sanitaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si l'impact économique de cette instruction a été appréhendé ou sera étudié prochainement par les services de votre ministère ? Combien de temps durera l'interdiction de la consommation de fromages au lait cru en restauration collective ? Envisagez-vous de la lever afin que ces produits, auxquels les Français sont attachés, puissent être exempts de soupçons

un syndrome hémolytique et urémique est 110 fois plus élevée. C'est la raison pour laquelle cette instruction a été donnée. Nous n'avons pas encore de retour d'expérience ; il y a de toute façon assez peu de fromages au lait cru,

en janvier dernier, vous déclariez que l'enseignement agricole était au coeur de vos priorités. C'est une ambition que nous ne pouvons que partager. Or, force est de constater que cette filière de formation, qui prépare à plus de deux cents métiers dans de nombreux domaines, demeure, hélas, peu attractive. À l'heure actuelle, l'enseignement agricole, qui est piloté par votre ministère, qui fait partie du service public de l'éducation, est bien le deuxième réseau éducatif français. À ce jour, ce sont 806 établissements répartis sur l'ensemble du territoire qui accueillent 160 000 élèves de la classe au brevet de technicien supérieur, chiffre auquel s'ajoutent quelque 35 000 apprentis. Quelque 40 % des formations proposées sont en lien avec la nature- agriculture, forêt, environnement, agroalimentaire, paysage, horticulture, viticulture -et ouvrent sur une très large gamme de métiers ou permettent d'intégrer l'enseignement supérieur agricole, qui, avec douze écoles publiques, délivre des diplômes de vétérinaire, d'ingénieur agronome, de paysagiste ou encore de professeur de l'enseignement agricole. Dernière précision, et non des moindres, l'enseignement agricole, très largement ouvert sur le monde, avec des échanges européens et internationaux Erasmus et la coopération, permet aux jeunes de trouver facilement un emploi au terme de leur scolarité. Aussi la confidentialité entourant cette filière est-elle d'autant plus incompréhensible. Ma question est donc simple : pourquoi, avec votre collègue de l'éducation nationale,

vous parlez d'or : l'enseignement agricole est un joyau, une pépite. Laissez-moi vous expliquer comment nous communiquons. Lorsque j'ai été nommé à mon poste, j'ai immédiatement

à tous les échelons, et singulièrement à celui de l'éducation et de la formation. J'entends votre réponse. Vous me dites que la courbe est inversée et que les effectifs sont désormais en hausse.

de certains équipements des jeux Olympiques de 2024, mais aussi sur les surcoûts, relevés en mars 2018 dans un rapport de l'inspection générale des finances

On évoque des offres qui se situeraient au moins entre 25 % et 30 % au-dessus du budget prévisionnel de 113 millions d'euros

est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, vous évoquez la question du centre aquatique et de la passerelle de Saint-Denis. Effectivement, nous devons veiller en permanence à ce que la construction des équipements entre dans les délais prévus pour une livraison

Aujourd'hui, la quasi-totalité du foncier nécessaire à l'accueil des sites olympiques a pu être sécurisée. La Solideo a avancé sur la sélection des prestataires

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les règles applicables en matière architecturale, notamment dans le périmètre de protection d'un bâtiment classé. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine avait pour objectif de conforter et de moderniser la protection des patrimoines en simplifiant le droit des espaces protégés, tout en rendant ce dernier plus intelligible pour les citoyens. Dans le cadre des débats organisés lors de l'élaboration de ce texte par la commission de la culture du Sénat, la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes convenait que « la loi, intelligemment, prévo[yait] désormais un périmètre réfléchi selon les perspectives et les abords d'un monument classé, au lieu des systématiques 500 mètres » et que « la loi port[ait] une ambition nouvelle pour la qualité architecturale. « nécessaire de marier l'architecture contemporaine et les sites classés ». Dans les faits, malheureusement, le traitement réalisé par les services des directions régionales des affaires culturelles et des unités départementales de l'architecture et du patrimoine ne va absolument pas dans ce sens. Sur le terrain, dans nos départements respectifs, le développement des communes, notamment rurales, est très largement contraint aujourd'hui en matière de consommation des espaces agricoles, avec un empilement de réglementations : PLU, SCOT, PLH, etc. etc. Que nous réserve l'avenir ? Nous n'avons qu'une seule certitude : les restrictions seront de plus en plus fortes et les contraintes encore plus grandes. Le Premier ministre a d'ailleurs déclaré au congrès de l'Association des maires ruraux de France, en 2019, que le Gouvernement souhaitait « lutter lutter contre l'artificialisation des sols, ce qui impliqu[ait] de renforcer les outils disponibles pour réhabiliter le bâti ancien ou pour mieux réguler les activités commerciales. » Il a ajouté : « Il faut faire attention au développement des espaces urbains ou périurbains ». Si les communes rurales et périurbaines veulent continuer d'être dynamiques, il faut permettre une réhabilitation du bâti existant, même dans les périmètres de protection d'un bâtiment classé. Sinon, des communes seront totalement privées de toute perspective d'évolution en matière architecturale. Aujourd'hui, les rejets des demandes de permis semblent beaucoup trop systématiques et bien souvent déconnectés des réalités locales. Il est indispensable de se donner les moyens de rénover et de moderniser de nombreuses habitations. On ne peut pas mettre des secteurs entiers de nos communes « sous cloche

est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur Bernard Fournier, la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, voulue par le Gouvernement, a introduit un nouveau dispositif de protection des abords de monuments historiques, que vous avez détaillé. L'objectif était de remplacer progressivement, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques par des périmètres délimités des abords (PDA), définis dans le code du patrimoine et plus adaptés à la réalité et aux enjeux locaux. de la loi, plus de 300 PDA de monuments historiques ont été institués. Les collectivités territoriales se sont bien approprié ce dispositif, qui tend à préserver un espace cohérent avec les monuments historiques qu'ils englobent. Notons que ces périmètres sont aussi validés après concertation avec la population, l'enquête publique. En leur sein, tous les travaux sont soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Les projets doivent concilier la préservation du patrimoine et la qualité architecturale du bâti, en tenant compte des enjeux d'habitabilité et de développement durable. L'un des objectifs est d'éviter l'étalement urbain et les évasions commerciales, dans le cadre du plan national « Action coeur de ville ». Nous pensons que le projet architectural contemporain de qualité participe de la démarche patrimoniale, de son dynamisme et de sa pérennité. Le patrimoine peut ainsi évoluer grâce à la création architecturale : il s'agit de réhabiliter des bâtiments en leur donnant une nouvelle fonction, en agrandissant des architectures existantes ou en s'y insérant. C'est l'un des enjeux de la lutte contre l'étalement urbain. Ainsi, l'architecture contemporaine a pu être introduite au sein de nombreux sites protégés au titre de code du patrimoine. Nous pouvons, notamment, citer les exemples du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Sedan, du musée des Beaux-arts de Dijon ou encore de l'école de musique de Louviers. comme a pu le dire le ministre de la culture à l'occasion des dernières Journées nationales de l'architecture : « Penser transformation et adaptation, [ ...] c'est sortir peu à peu de la logique du jetable au profit du recyclable et du réparable, sur le plan culturel comme sur le plan environnemental. »

Merci